les articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la régularisation d'étrangers par le travail. Cependant, les articles L. 8251-1 à L. 8256-8 du code du travail prévoient à l'encontre des employeurs recrutant des étrangers en situation irrégulière

n'est-il pas temps de faire évoluer ces règles en permettant un recrutement temporaire plus facile ? Cela permettrait de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et de contrôler plus facilement les étrangers non régularisés-

Elle doit également s'acquitter sous certaines conditions d'une taxe à payer dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de travail. Les employeurs sont donc tenus de se conformer à leurs obligations légales. Ils acceptent les risques, notamment pénaux, s'ils décident sciemment de contourner la réglementation. Il peut toutefois arriver que l'entreprise découvre que son salarié est étranger, qu'il a utilisé de faux documents d'identité ou qu'il a présenté un faux titre de séjour l'autorisant directement à travailler. Dans ce cas de figure, l'entreprise peut décider de licencier le salarié en question ou l'aider à obtenir sa régularisation auprès de la préfecture. Les travailleurs en situation irrégulière peuvent demander une admission exceptionnelle au séjour s'ils justifient

La circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, ne crée pas de droits opposables, mais énonce « des orientations générales destinées

des outre-mer. Madame la ministre, avec le réchauffement climatique, le risque d'incendie devrait malheureusement s'intensifier et s'étendre à l'ensemble du territoire national à l'avenir. C'est particulièrement vrai dans le département de la Nièvre, qui comporte de nombreux espaces forestiers, notamment

De ce point de vue, il est essentiel que les SDIS disposent des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de plus en plus complexes et nombreuses, et bien souvent extrêmement périlleuses. Le Gouvernement y est attentif, en lien avec les départements et les communes. Comme vous le savez, un agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative. Le cumul simultané de deux emplois publics permanents à temps complet est, en principe, interdit. Un fonctionnaire peut toutefois occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet. Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps non complet avec un emploi permanent à temps complet, en respectant toujours cette limite de 15 %.

et des outre-mer. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur la saturation des dispositifs de délivrance des titres d'identité. La délivrance d'un passeport ou d'une carte d'identité est devenue un véritable casse-tête pour les Français et pour les mairies. Dans le département du Bas-Rhin, certains délais avoisinent les six mois d'attente, auxquels il faut ajouter le temps d'instruction et de fabrication. En 2017, le Gouvernement réduisait considérablement le nombre de communes pouvant établir des titres d'identité. Aujourd'hui, le système est saturé, alors même qu'il s'agit d'une compétence dévolue à l'État ! Nous nous retrouvons face à un système « perdant-perdant

pour la ruralité ! Votre plan d'urgence, annoncé au mois de mai, a révélé le manque d'anticipation. Surtout, il s'avère insuffisant. La situation est toujours aussi difficile dans nos mairies. Je voudrais ici saluer le travail des élus locaux et des agents, qui agissent au mieux pour parvenir à répondre aux nombreuses demandes. Il faut davantage de lieux d'enregistrement. Il faut également équiper de nouvelles communes, ce qui limiterait les déplacements de nos concitoyens. Madame la ministre, il est nécessaire que les maires puissent disposer de moyens financiers et humains à la hauteur de cette mission, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il est urgent d'entendre les élus locaux et le mécontentement de nos concitoyens. Aussi, ma question est simple comment envisagez-vous de soutenir de manière pérenne les mairies et les élus locaux afin que cette mission de service public soit accessible à tous et puisse être exercée de nouveau efficacement, en tenant compte de la proximité

(ANTS) versera pour sa part une prime d'installation forfaitaire de 4 000 euros pour l'ouverture d'un centre temporaire et continuera de verser la prime d'installation de 4 000 euros qui accompagne tout déploiement d'un nouveau dispositif fixe à titre pérenne dans un nouveau site.

L'article L.O. 141 du code électoral précise que « le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris,

et un autre mandat local. Deuxièmement, au sein d'un même territoire métropolitain, des élus peuvent cumuler trois mandats et d'autres deux. À titre d'exemple, un parlementaire de la métropole peut être à la fois conseiller municipal et conseiller métropolitain, alors qu'un conseiller régional doit choisir entre son mandat de conseiller municipal métropolitain. S'il ne s'agit pas de commenter le bien-fondé de la limitation du cumul des mandats, je souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter une égalité entre tous les élus et faire ainsi entrer la métropole de Lyon dans le droit commun. La parole est

ne figure effectivement pas celui de conseiller de la métropole de Lyon. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi de ratification de l'ordonnance du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon que la nécessité d'une législation ultérieure avait été identifiée par les parlementaires. Cette ordonnance précisait les modalités d'élection des conseillers métropolitains, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi Maptam, qui a créé la métropole de Lyon.

Monsieur le ministre, au mois de juin dernier, j'interrogeais votre prédécesseur sur le nécessaire élargissement de la liste des produits concernés par le bouclier qualité-prix créé pour lutter contre la vie chère

Avec des prix à la consommation de 7 % à 13 % plus élevés que dans l'Hexagone, et des produits alimentaires plus chers de 19 % à 38 %, nos compatriotes d'outre-mer subissent de plein fouet l'inflation actuelle. C'est beaucoup pour des territoires dont vous n'ignorez pas les difficultés du point de vue de l'emploi et de la pauvreté. Lors de votre déplacement à la Réunion au début du mois de juillet, puis à l'Assemblée nationale, vous avez indiqué vouloir étendre le bouclier qualité-prix à « beaucoup plus de produits dont le prix serait bloqué, voire diminué

Les entreprises nationales et internationales, les grandes surfaces, les compagnies maritimes et les fournisseurs devraient ainsi se réunir à Paris pour trouver des solutions et s'entendre sur de nouveaux objectifs. Ma question est très simple : sans préjuger bien sûr des échanges qui se tiendront à la rentrée prochaine, pouvez-vous nous dire concrètement à quoi pourraient bien ressembler les prochains paniers du bouclier qualité-prix ? Le ministre Gérald Darmanin a par ailleurs précisé que les collectivités territoriales seraient associées aux discussions en raison de leur pouvoir d'action sur la fiscalité locale. Que pouvez-vous nous dire des pistes aujourd'hui à l'étude ? la lutte contre la vie chère est évidemment l'une des priorités du Gouvernement. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, nous connaissons actuellement une inflation mondiale inédite qui pèse plus encore sur les territoires ultramarins, non pas parce que l'inflation y augmente plus vite, mais parce qu'elle s'exerce

nous devons aller plus loin. C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu deux propositions que vous connaissez : la limitation de la hausse des loyers de référence à 2,5 % dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), contre 3,5 % dans l'Hexagone et le financement d'une aide supplémentaire de 15 millions d'euros pour prendre en compte le nombre élevé de nos concitoyens ultramarins modestes qui ne bénéficient pas des minima sociaux. J'ajoute que 4 millions d'euros ont été réservés aux territoires du Pacifique. Au-delà de ces mesures d'urgence, Gérald Darmanin et moi-même avons lancé l'initiative d'un Oudinot du pouvoir d'achat- je préfère cette dénomination à celle d'Oudinot de la vie chère.

territoriales. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur une question qui m'est remontée du terrain et qui concerne l'indemnisation des artistes en cas d'annulation d'un spectacle par la commune lorsqu'une tempête est annoncée. En effet, lorsqu'une commune passe commande auprès d'un groupe de musique pour la tenue d'un concert et que, le matin de l'événement, la préfecture relaye un bulletin d'alerte météorologique orange ou rouge, la municipalité décide alors d'annuler la représentation pour des raisons de sécurité. Plusieurs questions se posent alors. Si l'événement météorologique a effectivement lieu, le groupe est-il fondé à réclamer des indemnités à la commune ? Le cas échéant, celles-ci diffèrent-elles selon que l'événement a été qualifié, ou non, de cas de force majeure ? Si l'événement météorologique n'a finalement pas lieu, le groupe est-il tout de même fondé à réclamer des indemnités à la commune qui a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police au titre des informations reçues des services de l'État ou de Météo-France ? Existe-t-il un fonds gouvernemental pour indemniser les entrepreneurs de spectacle dans ces circonstances et, à défaut, est-il envisageable d'en créer un ? La La seule alerte orange ou rouge constitue-t-elle en elle-même un cas de force majeure, que l'événement météorologique ait finalement lieu ou non ?

? La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Détraigne, lorsque le spectacle est organisé par la commune, de telles conséquences n'engagent pas l'État, mais la seule commune ayant contracté avec le prestataire chargé de la représentation en cause. Dans cette hypothèse, les conséquences de l'annulation du spectacle sont régies par les stipulations contractuelles qui auront été prévues pour l'événement, notamment les conditions d'indemnisation. Dans le cas où l'événement météorologique n'aurait

Par ailleurs, un événement est qualifié de cas de force majeure en raison de son caractère imprévisible et irrésistible. En matière de marchés publics, cette hypothèse est prévue par l'article L. 2195-2 du code de la commande publique qui prévoit que ce motif justifie la résiliation du contrat par l'acheteur.

revanche, si le spectacle n'est pas organisé par la commune et que celle-ci met en oeuvre ses pouvoirs de police administrative pour l'interdire au regard des risques météorologiques, le prestataire de spectacle pourra chercher à mettre en cause la responsabilité de la commune. Celle-ci ne pourra être engagée que si une faute a été commise dans l'évaluation du risque météorologique. S'agissant des indemnités liées à l'annulation de la représentation, celles-ci seront déterminées par les clauses du contrat

L'objectif évident de préservation de la santé publique ne saurait être remis en cause, mais il me paraît important de rappeler que le principe de quotas fondés sur des critères démographiques, comme l'indique le code de la santé publique, est un héritage de mesures contre l'alcoolisme édictées dès 1955 dans le code des débits de boissons en vigueur à l'époque, lorsque le volume moyen de consommation d'alcool par Français excédait bien largement ce que nous connaissons aujourd'hui. Les évolutions de la société française, favorisées dans les années 1960 et 1970 par l'important exode rural, ainsi que par le passage d'une consommation annuelle de 200 litres d'alcool par Français en 1960 à moins de 80

Un assouplissement de cette règle serait pourtant largement bienvenu afin de permettre à des communes rurales de s'engager dans une démarche de revitalisation de leur territoire et de création de nouveaux lieux de convivialité, comme le promeut l'initiative Mille cafés, encouragée- entre autres -par le ministère de la cohésion des territoires.

Celles-ci ne seront toutefois pas transférables au-delà d'une même intercommunalité, afin d'éviter le départ de certains débits de boissons vers des territoires plus attractifs. Cette loi a également permis de revenir à un cadre départemental de gestion des licences, le passage en 2015 à un cadre régional ayant conduit à un transfert de trop nombreuses licences de zones fragiles économiquement vers des zones plus attractives. Enfin, la règle du seuil de population ne s'applique pas aux créations de licences de restaurants ni à celles des licences de vente à emporter, qui contribuent aussi à la vitalité de nos territoires.

quelles mesures réelles, pérennes et différenciées comptez-vous prendre pour les différents territoires d'outre-mer ? La

Concernant la Guadeloupe, la stratégie pauvreté a permis de financer la mise en place du SAMU social et son extension, en 2023, à toute la Guadeloupe continentale. Plus de quatre-vingts projets en faveur des publics précaires destinés à l'amélioration du logement et du cadre de vie, à l'accès à la culture, à la santé et à l'emploi ou encore à l'inclusion numérique ont été financés

Dans cet établissement, la diminution du nombre de lits d'hospitalisation, décidée ces dernières années, nuit à la qualité du service public rendu, comme j'ai pu le constater sur place. Les chiffres sont éloquents : plus de cinquante lits ont fermé depuis 2015 ; une unité est en cours de fermeture, soit dix-huit lits supprimés, et le futur projet d'établissement prévoit la fermeture de plusieurs unités d'admission. Face à cette réalité statistique, le personnel s'inquiète à juste titre du traitement réservé à certains patients, mais également d'une régulation forcée des admissions le week-end, ou encore de l'ajout de lits de camp en période de saturation. Les conséquences sont inquiétantes, tant pour les soignants qui essaient de trouver des places disponibles que pour les patients dont les pathologies, au sein de ce centre hospitalier, sont très spécifiques. Cette restructuration affaiblit considérablement l'offre de soins, l'accès aux soins, ainsi que la qualité de l'accueil et de la prise en charge par l'établissement. Au lendemain d'une crise sanitaire qui a mis en lumière les failles structurelles du système de soins hospitaliers, quelles mesures comptez-vous prendre, madame la ministre, pour que les restructurations internes à l'hôpital public, et plus particulièrement celui de l'hôpital psychiatrique La Candélie à Agen, ne riment pas avec suppressions de lits et baisse de la qualité des soins le centre hospitalier départemental (CHD) La Candélie est le seul établissement psychiatrique du département de Lot-et-Garonne. Comme beaucoup d'établissements spécialisés, il se caractérise par un nombre très important de patients atteints de maladies chroniques, dont la prise en charge relève avant tout de l'accompagnement médico-social. Aussi, progressivement, une évolution visant à réduire le nombre des unités accueillant des malades dits « chroniques » et à orienter ceux-ci vers une prise en charge médico-sociale a été privilégiée. Par ailleurs, dans le cadre du « virage ambulatoire », l'établissement a fermé plusieurs lits, afin de redéployer une partie de son activité vers des prises en charge externes, avec transfert de moyens au bénéfice de structures de type « centres médico-psychologiques » (CMP), hôpitaux de jour et équipes mobiles. Depuis 2015, les processus d'adaptation continus mis en oeuvre par le CHD et la diversification de ses activités ont conduit aux mesures suivantes : le 1 mars 2015, fermeture de l'unité des Acacias

mais, au moins, le CHD ne propose pas une nouvelle réduction de ses capacités par rapport à la situation actuelle.

et de la prévention. Madame la ministre, ma question porte sur la mise en oeuvre des dispositions du Ségur de la santé qui affiche, je le rappelle, l'ambition de fédérer les acteurs de santé dans les territoires autour de projets communs, censés être décloisonnés pour répondre au mieux aux besoins de la population. Il a été proposé de faire des hôpitaux de proximité de véritables laboratoires de la coopération territoriale dans le but de constituer un premier niveau de gradation des soins, en lien étroit avec les professionnels de ville, au sein notamment des communautés professionnelles territoriales de santé Le 21 décembre 2021, vingt-cinq établissements ont été labellisés par l'agence régionale de santé (ARS) sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont ceux de Gray, Lure et de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône.

J'en viens à ma question. Madame la ministre, en parfaite convergence de vue avec le maire de Luxeuil-les-Bains et l'ensemble des élus municipaux, je souhaiterais que vous me précisiez les mesures que afin de rouvrir en priorité, et dans les meilleurs délais possible, le service des consultations non programmées du site de Luxeuil-les-Bains, quatrième commune du département de la Haute-Saône.

de Passavant-la-Rochère à Faucogney-et-la-Mer, serait écartée encore plus durablement de l'organisation des services d'urgence, situation qui, comme vous l'imaginez, complique grandement l'installation de médecins généralistes. La parole est à Mme la ministre

Comme vous le mentionnez, trois sites du groupe hospitalier de la Haute-Saône, le GH 70, ont été labellisés « hôpitaux de proximité » à la fin de 2021. Cette labellisation traduit la dynamique et la volonté du groupe hospitalier de s'appuyer sur ces structures pour conforter son ancrage territorial, afin d'améliorer l'accès aux soins et le parcours des patients. Cette volonté se manifeste par la mise en oeuvre d'importants projets immobiliers financés dans le cadre du Ségur de la santé, qui visent notamment l'implantation de nouvelles unités sur chacun de ces sites. On peut citer à cet égard la création d'un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), d'une unité médicale post-urgence et le renforcement des consultations avancées de spécialité

l'objet de travaux de modernisation financés par des investissements du Ségur de la santé avec, pour objectif, au-delà du développement de l'activité d'hôpital de jour en médecine, du déploiement d'un SSR, d'un temps partiel et du renforcement des consultations avancées de spécialité, la réouverture du service des consultations non programmées (CNP) à Cette réouverture des CNP n'est envisageable que si se noue une collaboration étroite entre les praticiens hospitaliers et les médecins de ville pour assurer ensemble ce service. À ce titre, les médecins libéraux de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Luxeuil-les-Bains se mobilisent : un protocole de coopération et d'organisation est en cours d'élaboration entre la CPTS et l'hôpital. L'ARS de Bourgogne-Franche-Comté accompagne pleinement cette démarche. J'en profite pour souligner le dynamisme des CPTS au niveau national et leur rôle dans la coordination des acteurs sur les territoires et dans l'amélioration des parcours.

et de la prévention. Madame la ministre, la Mayenne comme de nombreux autres départements, connaît la crise des urgences, le manque de médecins généralistes et spécialistes. Les inégalités territoriales d'accès aux soins continuent de se creuser : 30 % des Français vivent aujourd'hui dans des territoires mal dotés ; près de 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins

comme l'hôpital Jules-Doitteau à Villaines-la-Juhel en Mayenne, souhaiteraient pouvoir prétendre à la labellisation, mais ne disposent pas d'une autorisation de médecine, qui est une des conditions requises par l'appel à labellisation. L'hôpital Jules-Doitteau ne fait donc partie ni des centres hospitaliers ni des hôpitaux de proximité, ce qui nuit aux professionnels, ainsi qu'à la population locale, et conduit à une perte d'identité dans le paysage sanitaire mayennais. Cet hôpital joue pourtant un rôle majeur de relais dans l'offre hospitalière départementale, en lien notamment avec le centre hospitalier du Nord-Mayenne et celui de Laval. La labellisation lui permettrait non seulement de retrouver une identité locale, mais aussi de prétendre à des moyens financiers supplémentaires. Aussi, je souhaiterais savoir, madame la ministre, si vous comptez élargir les labellisations « hôpital de proximité » aux établissements ne disposant pas d'une autorisation de médecine.

sous toutes ses formes, que ce soit sous la forme de maisons de santé, d'équipes de soins primaires ou de communautés professionnelles territoriales de santé. En cela, les hôpitaux de proximité ont vocation à constituer un réel trait d'union entre l'ensemble des acteurs libéraux, hospitaliers et médico-sociaux, pour proposer une offre de soins davantage structurée et des parcours plus fluides pour les usagers. Comme vous le rappelez, la labellisation relève d'une démarche volontaire des établissements de santé et aboutit à un nouveau modèle pour les hôpitaux que l'on peut qualifier de « laboratoire » en matière de coopération territoriale, des modes d'organisation ouverts sur leur territoire facilitant l'émergence d'organisations partagées et décloisonnées, des instances de pilotage et de décision élargies à des personnalités extérieures et un financement sécurisé. 24 juillet 2019 a défini le cadre de la labellisation, lequel précise le périmètre des activités obligatoires des hôpitaux de proximité : ces établissements exercent une activité de médecine, proposent des consultations, donnent accès à des plateaux techniques et à des équipements de télésanté. C'est l'engagement à remplir ces missions qui fonde le modèle de l'hôpital de proximité.

autre hôpital local. Ce rôle pivot en gériatrie se traduit par ailleurs par des coopérations ou une gouvernance partagée avec d'autres Ehpad sur le territoire. Cet hôpital n'a pu être labellisé comme « hôpital de proximité », car il ne dispose pas d'une autorisation d'activité de soins

d'eau par des adeptes du canyoning, entraînant une légitime inquiétude de leur part quant à la présence d'éléments dangereux pour la santé. Le maire de la commune d'Aiglun a fait réaliser des analyses par le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (Smiage) des Alpes-Maritimes, analyses qui ont révélé une pollution grave, due à la présence de bactéries d'origine fécale et de produits chimiques. Le maire a donc été obligé de prendre un arrêté pour interdire l'accès à la clue du Riolan à tous les usagers, qu'ils soient baigneurs ou pratiquants de sports en eau vive. Un important travail de concertation a été mené en parallèle par les communes d'Aiglun, de Sigale et l'agence régionale de santé,

afin de permettre aux maires de s'appuyer sur des normes précises pour protéger l'ensemble des populations qui ignorent les risques encourus ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, les sites de loisirs aquatiques sans activité de baignade, dans lesquels peuvent être pratiqués des sports d'eau vive, n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux eaux de baignade figurant aux articles L.

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE concerne les seules eaux de baignade, définies comme toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.

Une première proposition de nouvelle directive de la Commission européenne est attendue dès 2023 et pourrait faire évoluer la réglementation applicable en la matière dans les prochaines années. En attendant l'issue de ces travaux, il faut rappeler rappeler qu'il n'existe pas de réglementation sanitaire spécifique aux zones de loisirs nautiques sans activité de baignade. Les ARS ne sont ainsi pas compétentes pour mettre en oeuvre un contrôle sanitaire sur de tels sites. En revanche, elles le sont pour accompagner les acteurs locaux dans la caractérisation et l'évaluation de potentiels risques sanitaires, ainsi que la définition des mesures de gestion, y compris des recommandations sanitaires à mettre en oeuvre pour la protection du public. Si un risque pour la santé des personnes a été mis en évidence, des mesures de restriction et d'interdiction des sites peuvent être prononcées sur le fondement des pouvoirs de police municipale et de police préfectorale.

corrélé à la constante augmentation des attaques de troupeaux ces dernières années, nous ne pouvons pas rester sans réaction. Pour pallier les difficultés rencontrées par les éleveurs, nous avions, dès août 2020, adopté une résolution européenne visant à modifier le classement dont bénéficie le loup au sein de la convention de Berne. Malheureusement, aucune suite n'y a été donnée par le Gouvernement. de simplification de l'action publique locale, j'avais déposé un amendement qui prévoyait la possibilité de déroger au prélèvement défini au niveau national dans certaines zones où les attaques causent des dommages importants, en dépit de la mise en oeuvre de mesures de protection.

De même, je souhaiterais savoir si le Gouvernement compte revoir sa position quant à l'opportunité de créer des zones de protection renforcée contre les attaques de loups. Enfin, j'aimerais connaître, monsieur le ministre, votre position sur une éventuelle augmentation des moyens alloués à l'Office français de la biodiversité,

Imaginez, moins de 66 % des enseignements ont été dispensés au cours de l'année ! Cela représente une moyenne de dix heures d'absence par semaine, avec une tendance à l'augmentation qui n'a cessé de s'aggraver. Ce problème est loin d'être un cas isolé que ce soit en lycée professionnel, en lycée général, en collège ou même en primaire, ce constat est très largement partagé dans les établissements scolaires du département du Nord. Il s'agit d'absences nombreuses, fréquentes et prolongées que les écoles n'arrivent pas à combler, essentiellement par manque de moyens humains.

L'engagement de l'éducation nationale doit être sans faille et aucun enfant de la République ne peut en être privé. Madame la ministre, quelles sont les mesures mises en place par le Gouvernement pour corriger le remplacement insuffisant des enseignants et rétablir la continuité du service public pour tous les élèves

selon leurs spécialités ; je prendrai l'exemple de la santé au lycée Valentine-Labbé, de l'économie-gestion à la faculté de droit ou au lycée Gaston-Berger, ou encore à l'université polytechnique Hauts-de-France pour les filières industrielles et scientifiques. Plus généralement, nous avons mis en place un partenariat spécifique avec Pôle emploi, afin de bénéficier d'une source de recrutements supplémentaires, ainsi qu'un accompagnement des nouveaux contractuels par les corps d'inspection, et enfin des contrats de plus longue durée pour fidéliser ces contractuels. Au-delà du sujet des recrutements, nous sommes évidemment très engagés sur la question des remplacements, vous l'avez évoqué, madame la sénatrice. Cependant, la préoccupation principale du ministre de l'éducation nationale a trait évidemment à la continuité et à la qualité du service public. Pour cela, il est évident que chaque élève doit avoir un professeur en face de lui, pour l'ensemble de ses heures de cours, afin d'accompagner son cursus scolaire. Nous avons également

Recourir aux contractuels et aux étudiants, comme vous le proposez, ne fait que reporter la recherche d'une solution au problème. C'est une réponse conjoncturelle et pas une réponse structurelle. Plus on attend, plus les dégâts seront importants.

L'école tente d'y pourvoir. Alors que sa mission première est de transmettre les savoirs fondamentaux- lire, écrire et compter -et qu'elle donne à tous les élèves de France et de Navarre les outils nécessaires à la formation d'un esprit critique, l'école propose effectivement un éveil à la citoyenneté au moyen, parmi tous les apprentissages proposés, d'un enseignement moral et civique (EMC). Il est censé former et préparer les citoyens responsables de demain, les futurs électeurs.

que cette matière occupe une place par trop réduite dans les programmes scolaires, avec un volume horaire réservé aux cours d'EMC ne permettant pas d'étudier tout ce qui doit l'être. De plus, certains enseignants n'ont pas reçu de formation spécifique sur ce sujet. Quant au fonctionnement des institutions, il est quasiment absent des manuels scolaires.

est une mission fondamentale de l'école, doit être garantie à chaque élève. Pour cela, l'enseignement moral et civique tient une place prépondérante ; il est doté d'un volume horaire fixe et obligatoire du

public. Ces actions permettent à chaque acteur présent au sein de l'école de mettre en oeuvre cette mission fondamentale de l'éducation à la citoyenneté, qui est un facteur de réussite et d'épanouissement des élèves.

Madame la présidente, madame la ministre, les entreprises du secteur des logiciels, de l'ingénierie et de l'informatique payent une contribution obligatoire

je l'espère. La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous attirez l'attention du Gouvernement sur la contribution versée par les entreprises de la branche professionnelle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil

du 21 décembre 1999. Son maintien a été confirmé à plusieurs reprises, et encore dernièrement, par l'accord du 28 avril 2021, lui-même étendu par l'arrêté du 4 février 2022, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur. Le ministre chargé du travail a examiné la légalité de la mise en place de cette contribution et de son maintien, ainsi que celle de l'organisation et du fonctionnement de cette association, dans le cadre de la procédure d'extension des accords collectifs. Je vous le rappelle : cette procédure a pour objet de rendre un accord collectif applicable aux entreprises non adhérentes ; il ne lui appartient en aucune façon de se prononcer sur l'opportunité des mesures adoptées par les partenaires sociaux. Le maintien de cette contribution et le fonctionnement de l'Adesatt concernent les entreprises et les salariés de la branche ; seul un nouvel accord de branche pourrait donc décider de son éventuelle suppression. J'attire toutefois votre attention sur le fait que cette contribution vise essentiellement à financer les actions liées au paritarisme. En 2021, près de 90 % des fonds collectés étaient affectés au soutien du paritarisme et favorisaient la diffusion ainsi que l'appropriation, auprès des entreprises et des salariés, des accords signés et des dispositifs mis en place, par exemple en matière de formation professionnelle ou de prévoyance.

vous interroger sur l'application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger. Cet article dispose que « l'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement ». Cela signifie,, que seuls les agents affectés à une mission auprès d'un ambassadeur seraient concernés, et non ceux qui exercent un autre emploi à l'étranger et ne dépendent pas hiérarchiquement de l'ambassadeur. « rappel de tout agent » laisse entendre que celui-ci serait rappelé auprès de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. De plus, le critère d'urgence n'est pas défini et semble être laissé à l'appréciation de l'ambassadeur. Enfin, on ignore si l'ordre de partir immédiatement concerne le fait de quitter l'emploi occupé par l'agent ou bien le pays étranger où l'agent exerce ses fonctions. Or cet article a servi de fondement à un ambassadeur pour intimer l'ordre de quitter l'emploi et le pays où il exerçait au directeur d'un établissement scolaire homologué de l'enseignement français à l'étranger. Cet établissement est géré par une association de gestion de droit local, qui était l'employeur du directeur d'établissement ; ce directeur était donc un fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale auprès d'un établissement d'enseignement français à l'étranger, homologué et relevant du droit local, et non un agent du poste diplomatique ou un enseignant détaché auprès de l'agence. L'ambassadeur n'était donc pas ici l'autorité compétente en matière disciplinaire. Cette demande de l'ambassadeur a eu pour conséquence directe le licenciement du directeur de l'établissement par l'association de gestion de l'école. Aussi, je vous demande de préciser les contours de l'application de l'article 9 du décret précité et, en particulier, de m'indiquer si, d'une part, cet article permet à l'ambassadeur d'exiger le départ d'un tel agent de son emploi et de son pays de résidence et, d'autre part, si un ambassadeur peut en faire application lorsque le fonctionnaire détaché est un salarié de droit local.

En vertu de l'article 1 du décret n° 79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, l'ambassadeur représente le Gouvernement et chacun des ministres. Les pouvoirs conférés aux ambassadeurs à l'article 9 du décret du 1 juin 1979, que vous citez, ne le sont pas en vertu de leur pouvoir disciplinaire propre, mais plus généralement en leur qualité de représentant du Gouvernement et de chacun des ministres à l'étranger.

signalements de crimes et délits, en complément des plaintes déposées par les victimes. L'établissement scolaire figurait dans la liste des établissements homologués pour l'année scolaire 2020-2021 définie par l'arrêté du 25 mai 2020 fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués. Les personnels de cet établissement ayant la qualité de fonctionnaire restent, dans l'exercice de leur mission, placés sous l'autorité du ministère ; ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'un rappel au titre de l'article 9. La parole est à Mme Patricia Demas, auteure de la

La Commission européenne retient néanmoins, pour les ZTD, un horizon temporel de trois ans afin d'estimer la probabilité d'une carence de l'offre privée et la possibilité d'une intervention publique, en lieu et place de l'opérateur d'infrastructures défaillant. Concrètement, cette carence est difficile à constater et la réponse apportée par la collectivité a peu de chance d'être de nature à satisfaire les usagers concernés, compte tenu de la durée et du coût nécessaires au déploiement des prises manquantes.

Permettez-moi, tout d'abord, de saluer le travail conjoint de l'ensemble des acteurs économiques, des élus locaux, des parlementaires et des collectivités locales, y compris dans votre département des Alpes-Maritimes, qui permet à la France, au sein de l'Union européenne, de figurer en première place s'agissant du déploiement de la fibre. En effet, en moins de dix ans de déploiement, 72 % des locaux sont éligibles à une offre fibre et plus de 80 % le sont à une offre très haut débit au moyen d'une technologie filaire. Le plan France Très Haut Débit, lancé en 2013, vise un déploiement du très haut débit pour tous nos concitoyens, vous l'avez rappelé. Pour atteindre cet objectif, et au regard du régime notifié en vigueur pour ce plan, que conformément aux règles d'attribution en matière d'aides d'État, les subventions sont mobilisées seulement sur la zone moins dense du territoire où la carence de l'initiative privée est établie. Sur les 20 milliards d'euros d'investissements effectués en dix ans, plus de 3,3 milliards d'euros sont du ressort de l'État.

à proximité des logements situés dans ces zones de forte densité. Une évolution législative, comme vous le suggérez, visant à renforcer cette recommandation de complétude pourrait soulever des questions relatives à la prévisibilité et à la stabilité du cadre législatif et réglementaire du déploiement de la fibre en France,

Cela dit, je peux vous assurer que le Gouvernement et mon ministère sont pleinement mobilisés sur ce sujet et travaillent avec l'Arcep afin d'assurer l'accès au très haut débit à l'ensemble de nos concitoyens.

Comme vous le savez, plus de 200 collectivités haut-rhinoises ont adopté une délibération contre ce texte et 130 d'entre elles ont engagé un recours afin que certaines adaptations soient envisagées pour tenir compte des spécificités de notre territoire, notamment des aménagements hydrauliques et des digues préexistantes. Vous le savez, le Haut-Rhin est un département pionnier s'agissant de la reconquête des zones inondables et de la biodiversité, ainsi que de la rétention des crues, puisqu'il est pourvu de plus de 200 kilomètres de digues et de près d'une centaine d'ouvrages qui contribuent à sa protection. Malheureusement, tel qu'il est envisagé chez nous, ce plan va à l'encontre des objectifs de la réglementation nationale et empêchera la construction de nouveaux bassins de stockage, ce qui laissera de nombreuses communes exposées aux coulées de boues et aux inondations. Il ne s'agit pas de remettre en cause les principes généraux du PGRI, ni d'ouvrir de nouvelles zones d'urbanisation, mais bien d'éviter que certains territoires ne soient « gelés » par des « espaces de précaution » placés en aval de ces ouvrages, des espaces déjà urbanisés, alors que les ouvrages derrière lesquels ils sont situés ont été conçus et validés par l'État pour résister à des épisodes centennaux et que, à ce titre, ils devraient être classés en zone jaune. Les élus haut-rhinois sont, par ailleurs, inquiets de voir une nouvelle compétence de l'État leur échoir, sans que les charges induites à venir soient compensées. Madame la ministre, le PGRI du bassin Rhin-Meuse est le seul en France à traiter de façon aussi restrictive les aménagements hydrauliques.

qui, ne pouvant être présent, m'a demandé de le représenter. Les PGRI sont élaborés dans chaque bassin de notre territoire et leur objectif, comme vous le savez, est de nous préparer aux risques d'inondation, qui vont être renforcés par les effets du changement climatique. Votre question porte sur les orientations prises dans le cadre du PGRI du bassin Rhin-Meuse, mais ces orientations sont, en réalité, les mêmes pour l'ensemble du territoire. En effet, les digues et les ouvrages ralentisseurs de crues

en un temps donné, s'affaiblissent au fil des années et deviennent incapables de retenir des crues, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un entretien rigoureux pendant des décennies. De plus, des ouvrages pensés

À l'inverse, toute implantation d'habitation nous engage pour plusieurs décennies et ces territoires ne sont que très rarement rendus à la nature ensuite. C'est la raison pour laquelle, depuis les années 1990, il est prévu une bande de sécurité afin de tenir compte de l'éventuelle défaillance des digues et des ouvrages ralentisseurs de crues. Cette orientation a d'ailleurs pris une valeur réglementaire en 2019 dans le décret encadrant les plans de prévention des risques d'inondation. Ce décret avait été élaboré en association étroite avec les collectivités, qui avaient d'ailleurs rendu un avis favorable à l'unanimité, lors de son examen par le Conseil national d'évaluation des normes. Les services du ministère dans la région

qui subiront une forte dévalorisation de leurs biens. Je voudrais rappeler que tous les ouvrages haut-rhinois ont été conçus et validés par l'État- c'est important -et nous regrettons que l'administration ne tienne pas compte de notre spécificité et fasse fi de l'avis de plus de 1 500 élus locaux, qui demandent à être écoutés. La parole est

Elle reçoit des subventions privées, notamment de la part de l'opérateur éolien Valorem, sa fondation Watt for Change, et de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), ce qui se conçoit aisément. cette association fait également état de subventions provenant du gestionnaire du réseau français de transport d'électricité (RTE), ainsi que de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). je souhaite connaître les motifs d'intérêt général qui justifient l'attribution de telles subventions par un établissement public et un organisme investi de missions de service public tels que l'Ademe et RTE. Par ailleurs, êtes-vous à même de garantir l'absence de conflit d'intérêts s'agissant de parcours professionnels qui passeraient de postes de direction dans le secteur des énergies renouvelables à des postes clefs à RTE ou à l'Ademe et singulièrement, bien sûr, à la commission d'attribution des aides ? La parole

conventions de financement et prévoient notamment la production de livrables. Il s'agit de projets précis, comme le développement d'un outil de modélisation de l'évolution de la production industrielle, la réalisation d'un projet de prospective de transition énergétique pour l'Europe ou ou encore la mise en place d'une application web pour structurer et piloter une trajectoire 2021-2050 de performance énergétique du bâtiment. S'agissant des modalités d'attribution des aides, l'Ademe applique les règles fixées par son conseil d'administration. En outre, elle suit une comitologie qui assure la transparence des prises de décision. En particulier, une personne ayant un intérêt dans un projet ne peut en aucun cas prendre part à une décision concernant ce projet. Lors des recrutements, la question de possibles conflits conflits d'intérêts est, elle aussi, examinée attentivement. J'en viens maintenant à RTE. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une entreprise investie de missions de service public. En tant qu'entreprise, RTE est libre de sa politique de mécénat et de partenariat. Cette politique comprend des partenariats très ciblés et limités dans le temps avec des organisations non gouvernementales (ONG) investies dans la transition énergétique. Ces partenariats ne portent pas sur les filières de production d'énergie. Ils sont conclus avec diverses organisations

techniques et opérationnels de l'activité de gestionnaire de réseau public de transport d'électricité. De nombreux salariés ont accumulé une expérience professionnelle dans le secteur de l'énergie préalablement à leur embauche

Le recours à des conventions de financement avec négaWatt peut paraître opportun. Néanmoins, on peut s'interroger quand on on constate la légèreté des orientations antinucléaires de la politique énergétique menée ces dernières années et les conséquences auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, avec la réouverture de centrales à charbon. La parole

En effet, de nombreux emplacements prévus pour la recharge des batteries des véhicules électriques sont monopolisés par des utilisateurs de véhicules électriques qui prolongent leur stationnement bien au-delà de ce dont ils ont besoin pour recharger leur voiture. Ce stationnement prolongé limite considérablement la rotation sur ces places. Un tel comportement abusif complique la possibilité de recharge pour nombre d'utilisateurs. De surcroît, ce phénomène ne peut que décourager les automobilistes de délaisser les véhicules thermiques au profit des véhicules électriques, étant donné qu'ils ne peuvent recharger leurs batteries dans des conditions acceptables. acceptables. L'article L. 417-1 du code de la route dispose que les véhicules stationnant en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière. fourrière. L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales précise quant à lui que le maire peut, par arrêté motivé, réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. J'ai été alerté par des élus locaux sur ce sujet : que faut-il faire pour lutter contre ce phénomène de « voitures ventouses » ? Pouvez-vous m'assurer que les dispositions légales citées s'appliquent bien aux véhicules électriques ? Sur quels dispositifs les maires peuvent-ils s'appuyer pour trouver des solutions efficaces ? On ne peut considérer que le délai de sept jours, nécessaire pour qualifier un stationnement d'abusif, soit pertinent pour les places destinées à la recharge. Le législateur ne devrait-il pas intervenir dans ce domaine, peu réglementé et pourtant crucial pour la transition écologique ? La parole est

et de la protection de l'environnement, le maire peut ainsi réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. Il peut également réserver des emplacements de stationnement aménagés, notamment aux véhicules à très faibles émissions au sens du code de la route : les véhicules électriques En outre, le maire dispose de la faculté de limiter la durée du stationnement pour tout ou partie de l'agglomération. En particulier, il peut imposer aux conducteurs de véhicules d'apposer sur ces derniers un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, par exemple un disque de stationnement. En toute hypothèse, si le code de la route définit comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, le maire peut tout à fait fixer, par arrêté, une durée inférieure. Un stationnement qualifié d'abusif est également puni de l'amende de 35 euros prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'ensemble des pouvoirs dont dispose le maire lui permet donc de favoriser la rotation des véhicules sur les places de stationnement, notamment sur les emplacements destinés à la recharge

des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales gestionnaires de la compétence assainissement sont confrontées à la problématique de la gestion des boues des stations d'épuration, particulièrement à la question de l'hygiénisation des boues.

En effet, dans le contexte de la crise sanitaire, plusieurs arrêtés portant sur la gestion des boues d'épuration urbaine ont créé de nouvelles contraintes pour les services d'assainissement des collectivités territoriales, comme l'impossibilité de l'épandage agricole pour les boues liquides non hygiénisées. Or les collectivités doivent avoir la visibilité nécessaire pour s'adapter aux modifications réglementaires à venir, relatives aux systèmes de traitement des boues, notamment pour répondre aux futurs critères d'innocuité et évoluer vers la siccité qui pourrait être requise.

quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour accompagner les collectivités dans la mise en conformité de la gestion des boues des stations d'épuration, et selon quel calendrier ? La parole

La gestion durable des boues de stations d'épuration est essentielle au bon fonctionnement de ces infrastructures et donc à la protection des milieux aquatiques, des zones de baignade ou encore, par exemple, de la conchyliculture. La réglementation encadrant l'épandage des boues date de 1998 : les nouvelles connaissances scientifiques et techniques acquises depuis lors justifient de renforcer les exigences de qualité des boues d'épuration destinées à une valorisation agronomique en agriculture. d'accroître ces exigences pour mieux protéger les sols, mieux protéger la ressource en eau et maintenir une relation de confiance entre les producteurs de boues, les exploitants agricoles et les consommateurs.

et donc leur valorisation. Par ailleurs, le Gouvernement vient de saisir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) pour obtenir une analyse du risque sanitaire, au regard de l'épidémie et des restrictions actuelles. Les discussions sur les projets de textes fixant le futur socle commun d'innocuité aux matières fertilisantes

préoccupations. Pour répondre à ces nouveaux référentiels, il nous faudra améliorer la qualité des boues. La priorité est de diminuer certaines pollutions rejetées dans les réseaux d'assainissement, effluents d'activités industrielles et artisanales

et rendre visibles les conditions de vie indignes d'une centaine de familles aujourd'hui à la rue ou mal logées. Ces familles comptent parfois de très jeunes enfants, dont certains handicapés et d'autres en mauvais état de santé. Elles sont en situation de grande précarité et peinent à se nourrir chaque jour. Alors que la chaleur et la sécheresse rendent la vie à la rue encore plus rude, les appels au 115 se révèlent souvent infructueux ; et, lorsque des hébergements sont proposés, ils sont très souvent inadaptés, accordés à titre temporaire et généralement très éloignés des écoles et des administrations. Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. L'inconditionnalité de l'accueil est en effet un principe inscrit dans le code de l'action sociale et des familles. De plus, nombre de ces personnes remplissent les critères permettant d'établir le caractère prioritaire de leur dossier au titre Or, depuis des années, des associations, des citoyens et des collectivités territoriales pallient les défaillances de l'État. À Grenoble, la ville a trouvé un hébergement pour ces familles pour le mois d'août et travaille à la réquisition de logements vacants. En Isère, on recense ainsi plus de 17 000 logements vacants et 3 300 bâtiments publics inoccupés.

Madame la secrétaire d'État, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour répondre à l'insuffisance actuelle des solutions de mise à l'abri et améliorer les conditions de vie dans les centres d'hébergement d'urgence ? Plus spécifiquement, quels moyens apportera-t-on en Isère pour répondre à la situation de ces dizaines de familles à la rue ? La

C'est d'abord une politique de prévention, pour agir en amont et limiter au maximum les discontinuités dans les trajectoires de vie. Des consignes ont ainsi été transmises aux préfets à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer le relogement de toutes les personnes qui feraient l'objet d'un concours de la force publique à l'issue de la trêve hivernale ou, à défaut, de leur proposer une solution d'hébergement et d'accompagnement adaptée à leurs besoins. C'est aussi une politique d'action pour toutes les personnes contraintes de recourir à l'hébergement d'urgence. L'État a ainsi fait de la politique du « Logement d'abord » le cadre de référence de son action de lutte contre le sans-abrisme depuis 2017, pour que les personnes hébergées accèdent le plus rapidement possible à un logement. Cette politique porte ses fruits : plus de 330 000 personnes sans domicile ont accédé au logement depuis 2018. Dans votre département de l'Isère, 1 269 personnes ont accédé au logement social au cours de la seule année 2021, grâce à l'implication constante de l'ensemble des acteurs. C'est enfin le financement d'un parc d'hébergements destinés à l'accueil inconditionnel des personnes ayant besoin d'être hébergées, principe fondamental ancré dans la loi française. Ce parc atteint aujourd'hui un niveau historiquement élevé : il dépasse désormais les 190 000 places, ce qui représente 20 000 places de plus qu'avant la crise sanitaire. En outre, l'État veille à ce que cette politique soit assortie d'un accompagnement de qualité pour chacun,

particulièrement vrai en Isère. Leur implication et leur dévouement, qui sont indispensables, permettent d'aboutir à des solutions concrètes. De même, il est indispensable que les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes, prennent pleinement leur part de responsabilité en lien avec les services de l'État pour répondre au mieux à ces besoins.